La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été mis en ligne sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

amorce le débat que nous allons avoir sur l'annulation des charges fiscales et sociales, qui mobilise mon groupe depuis

de nombreuses activités. Or le report de charges, à nos yeux, n'est pas pertinent. On ne peut pas demander à des gens qui ne vont pas percevoir de recettes pendant des semaines et des mois, qui ne savent pas quand ils vont pouvoir recommencer à travailler ni avec quels débouchés, de payer des taxes et des charges,

publiquement que les métiers de la restauration et de l'hôtellerie étaient prioritaires- personne n'en disconvient -et qu'on pourrait étudier au cas par cas

des charges fiscales et sociales.

Cet amendement vise à interdire en 2020 le versement de dividendes aux sociétés ayant bénéficié de la solidarité nationale dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Au regard de la gravité de la situation économique et de la mobilisation massive de la puissance publique, le ministre de l'économie et des finances a demandé aux entreprises qui bénéficient d'aides publiques- garantie, chômage partiel, fonds d'indemnisation -de renoncer au versement de dividendes en 2020. À ce stade, cette demande relève de la seule intention. Aussi cet amendement vise-t-il à inscrire dans la loi l'engagement demandé par le ministre de l'économie et des finances aux entreprises concernées. objet d'interdire en 2020 le versement de dividendes aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ayant bénéficié d'au moins une des aides directes ou indirectes de l'État mises en oeuvre pour amortir les effets économiques de la crise. Ne sont concernées que les sociétés dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions d'euros. Il s'agit d'exclure les petites entreprises, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ou les GAEC par exemple, afin de ne pas décourager l'actionnariat populaire. Cette interdiction s'étend à toute forme de dividende, y compris les avances et les intérêts sur premier dividende, qu'ils soient en numéraire ou en actions.

nous proposons s'inspire des mesures votées dans le cadre de la souscription nationale lancée en 2019 pour les travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris : il s'agit de porter à 75 % le taux de déduction d'impôts pour les entreprises, au lieu de 60 % actuellement. L'augmentation de cette déduction fiscale n'a pour seul objectif que de permettre de nouvelles sources de financement dans la durée pour accompagner la reprise économique post-crise et ainsi consolider notre réseau de petites entreprises, où travaillent un très grand nombre de salariés non délocalisables et qui participent à la richesse de nos territoires. Les fonds ainsi collectés seront réinvestis localement et viendront s'ajouter à la solidarité nationale engagée par l'État. Quel

Vall, est ainsi libellé : La parole est à Mme Nathalie Delattre. Le code du travail permet aux établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l'activité ou des besoins du public de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. période d'état d'urgence sanitaire, le rythme hebdomadaire de nos semaines de travail a été bouleversé. Pour de nombreuses chaînes de production, d'acheminement, de distribution et de vente, les jours se suivent

il est de notre devoir de leur dire merci avant de penser, demain, à une revalorisation sociale et financière de leurs métiers, lorsque nous serons sortis de la crise. Dans les commerces de détail alimentaires, en grande surface notamment, les salariés peuvent bénéficier d'une majoration de salaire pour le travail du dimanche. Cet amendement vise à encourager cette pratique en défiscalisant les éventuelles majorations de rémunération dominicale. Pour saluer le travail fourni sans relâche par ces Français sur cette ligne de front, je vous encourage, mes chers collègues, à adopter cet amendement. Quel

amendement a pour objet de clarifier et de corriger la rédaction de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en précisant son ciblage sur les loyers afférents à des immeubles loués par des entreprises, quelle que soit leur forme.

Cet amendement a pour objet de proposer une exonération fiscale et sociale totale de l'ensemble des heures supplémentaires travaillées pendant l'état d'urgence sanitaire, afin de soutenir les salariés particulièrement mobilisés. Les heures supplémentaires seraient exonérées d'impôt sur le revenu au-delà du seuil de 5 000 euros, ainsi que de cotisations patronales. Cet amendement constitue un complément utile à l'ordonnance du 1 avril 2020,

ligne : les soignants, les caissières de supermarché, des quantités de professions qui permettent à la France de tourner. La défiscalisation des heures supplémentaires est le moyen concret

Comme quoi, on peut être de droite et avoir des idées généreuses et de la morale. L'idée est extrêmement simple : pas d'aide pour les sociétés ayant un établissement ou une filiale dans un paradis fiscal.

que vous avez bien voulu voter précédemment et qui vient clarifier la rédaction de l'article adopté par l'Assemblée nationale sur la déduction fiscale et la neutralité fiscale

Monsieur le rapporteur

204. La commission des finances

Toutefois, elles n'auront que peu d'effets si vous ne clarifiez pas les conditions sanitaires et juridiques de la reprise. Cette crise n'est pas une crise économique classique, elle est à la base sanitaire. Si nous ne sécurisons pas plus clairement les chefs d'entreprise en leur indiquant jusqu'où va leur responsabilité vis-à-vis de leurs salariés en matière sanitaire, nous créerons une incertitude qui constituera, pour eux comme pour les salariés, un frein majeur à la reprise. Aujourd'hui, la situation n'est pas claire : le code du travail parle d'obligation de moyens, mais la jurisprudence oscille entre obligation de résultat et obligation de moyens. Les inspections du travail ont leur interprétation,

jusqu'où peut-on imputer à un chef d'entreprise la diffusion de l'épidémie parmi ses salariés ? Jusqu'où va précisément sa responsabilité en matière de fourniture de masques, de gants, de blouses ? Ce sont à ces questions, qui ont trait à la confiance, qu'il faut répondre avec précision.

les conditions de la reprise dépendront moins des tombereaux de milliards d'euros que nous déverserons sur l'économie que de la confiance que nous pourrons recréer.

la loi dispose que le chef d'entreprise a uniquement une obligation de moyens. Elle n'a pas tort, mais elle n'a pas non plus raison, puisque la construction prétorienne des tribunaux est telle le juge considère que le chef d'entreprise a le plus souvent une obligation non pas de moyens, mais de résultat. Il est absolument fondamental de trancher ce point pour que l'activité puisse reprendre.

le conflit entre ce que le législateur a prévu dans la loi et ce que la jurisprudence a inscrit dans cette construction prétorienne du droit social

de déconfinement, pour prendre cette expression, nous permettra, selon les délais proposés par le Président de la République, d'aborder ces sujets. Je note vos interventions et celles des autres parlementaires sur ce sujet comme autant de contributions et d'alertes. C'est un point d'attention que nous partageons et sur lequel nous allons nous pencher dans les jours qui viennent.

aux biens de protection de la personne dans une période de crise épidémique ne constituerait pas un gros écart par rapport au droit de l'Union européenne. Et si le Gouvernement présente une demande d'extension à cet objet

J'ai bien entendu les propos d'Alain Richard, mais l'honnêteté me conduit à dire que nous faisons déjà une interprétation assez large de la notion de produits médicaux

nous concentrer sur les cotisations patronales, le dispositif de chômage partiel permettant aux entreprises d'être dispensées du paiement des cotisations salariales pendant cette période, et trouver un dispositif conforme au droit communautaire.

de la construction. La profession est confrontée à une pénurie de main-d'oeuvre, au doute et à des difficultés liées à l'approvisionnement et à l'acheminement des matériaux. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique estime que 90 % des chantiers de rénovation Or la rénovation énergétique constitue l'un des piliers de la politique énergétique et climatique. Le secteur du bâtiment représentant 20 % de nos émissions nationales de gaz à effet de serre, il est indispensable de promouvoir les opérations de rénovation énergétique pour atteindre un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Le législateur a d'ailleurs prévu que 500 000 rénovations de logements soient effectuées chaque année, dont la moitié à l'attention des ménages modestes, dans le but de disposer d'un parc aux normes « bâtiment basse consommation » d'ici à 2050.

qui encadre l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % afférent aux travaux d'amélioration de leur qualité énergétique. C'est une mesure d'urgence qui doit permettre de répondre à la crise tout en favorisant l'atteinte effective des objectifs de notre politique énergétique et climatique. Quel est l'avis de la

Les acteurs économiques nous ont fait part de leurs demandes, que je souhaite ici appuyer : gel des redevances domaniales, exonération des taxes portuaires et paiement immédiat des indemnités d'assurance pour les sinistres existants avant la crise.

également l'intégration des pertes financières résultant d'une immobilisation des navires face aux risques sanitaires et à la pandémie dans la catégorie des risques de guerre, une intervention de la Caisse centrale de réassurance de l'État

qui ont constitué une déduction pour aléas (DPA) d'utiliser les sommes ainsi déduites et les intérêts capitalisés correspondants pour faire face aux dépenses nécessitées par l'activité professionnelle sans autre condition

le barème du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2020, le Sénat avait fait part de profondes réserves sur la transformation du CITE

des chaudières à très haute performance énergétique- avec quelques réserves -et la revalorisation de la prise en charge des poêles et cuisinières à bois dans un souci de

ainsi libellé : La parole est à M. Joël Labbé. Le présent amendement vise à permettre aux étudiants ayant contracté un emprunt auprès des banques pour le financement de leurs études de demander un report de leurs mensualités pendant la durée de la crise sanitaire.

contracté des prêts aux fins de pouvoir suivre un enseignement professionnalisant, sont à présent dans l'angoisse de ne plus être en mesure de les rembourser à temps. En effet, avec la mise en place du confinement, une grande partie d'entre eux a perdu le stage ou le travail étudiant qui leur permettait de faire face à ces dépenses. À cette exigence de remboursement s'ajoutent de nombreuses autres dépenses auxquelles doivent faire face les étudiants, pour leur logement, qu'ils ont dû garder, et leur approvisionnement alimentaire. La précarité étudiante n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui, et les difficultés financières risquent de se faire ressentir sur le long terme, car une part importante des 700 000 jeunes qui finissent leur formation initiale risque de se retrouver sans emploi face à la crise économique à laquelle nous devons faire face. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour ces étudiants si l'on ne veut pas creuser plus encore les inégalités entre eux. Tel est l'objet de cet amendement.

faire face à l'épidémie de Covid-19 permet aux microentreprises éligibles au fonds de solidarité de bénéficier de reports de paiement de leurs factures d'eau, d'électricité ou de gaz auprès de leurs fournisseurs.

50 % pour l'électricité par rapport à l'Arenh et 40 % pour le gaz par rapport aux tarifs d'il y a un an. Certains fournisseurs sont d'ailleurs contraints de revoir leurs grands investissements. À titre d'exemple, EDF a indiqué procéder à la remise à plat de son programme d'arrêts de tranche, c'est-à-dire d'opérations de maintenance du parc nucléaire existant. S'il est utile et nécessaire que les énergéticiens jouent sur leur trésorerie pour offrir de la souplesse aux microentreprises, je pense qu'ils n'ont pas vocation à prendre en charge d'éventuels impayés de facturation, ce qui dégraderait davantage encore leur situation financière déjà heurtée de plein fouet par la crise économique, qui est aussi une crise énergétique. énergétique. La solidarité nationale doit jouer. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet d'instituer un mécanisme de déduction d'impôt sur les sociétés pour les fournisseurs d'électricité, de gaz ou d'eau visant à compenser le montant des factures des microentreprises demeurant impayées à l'issue de l'application des reports de paiement.

arrêtée ou ralentie fortement pendant cette crise sanitaire. Certes, le Gouvernement a décidé un report des cotisations sociales et fiscales pour la période concernée. Néanmoins, ce choix

les acquitter. Or, dans la période que nous traversons, nombre d'entreprises voient ce chiffre d'affaires baisser drastiquement, jusqu'à devenir nul pour certaines. C'est pourquoi le report de ces cotisations ne réglera en rien les difficultés rencontrées, les ressources nécessaires à leur paiement n'ayant pas

Pour ces entreprises, nous souhaitons tout simplement une clarification. Nous voulons d'ores et déjà annoncer que les reports de charges se transformeront, de fait, en annulations de charges. Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à créer un crédit d'impôt et de charges

La liberté de la presse, valeur consubstantielle à notre démocratie, ne peut être garantie que par l'indépendance politique des organes. Cette indépendance, nous la devons à la capacité des entreprises de presse de ne pas vivre exclusivement des subsides publics, que ce soit au travers de l'aide directe de l'État à la presse ou des différents soutiens budgétaires assurés par les collectivités territoriales. Cette capacité, au-delà des ventes de papier, qui sont tendanciellement en chute, provient de la publicité.

peuvent être suspendus. Néanmoins, il ne s'agit que d'un report de ces échéances, qui ne suffira pas, même à court terme, car les pertes ne seront pas compensées à la sortie de la crise. Cet amendement vise donc à annuler, pour l'exercice comptable en cours, les impôts sur le revenu et sur les sociétés des exploitants et sociétés agricoles et viticoles. ces prélèvements étant calculés sur le fondement du ou des derniers exercices comptables, pour lesquels la situation économique était très différente, les maintenir serait fatal

Cet amendement est très sympathique, mais il vise à exonérer d'impôt sur le revenu l'ensemble des entreprises agricoles, ce qui est malheureusement anticonstitutionnel, car cela poserait un problème de rupture d'égalité devant les charges publiques. Je pense qu'il s'agit plus d'une position de principe ou d'un amendement d'appel

des tourteaux et des drêches, qui contribuent à notre indépendance protéinique, dont nous parlons depuis longtemps. Ainsi, vu les difficultés traversées par le secteur des biocarburants, mais aussi son intérêt économique et social avéré,

Parmi elles, la filière des huiles et protéines végétales a continué de produire des tourteaux de colza pour la nutrition de l'élevage animal, de l'huile alimentaire pour nos ménages et de la glycérine pour la production de gels hydroalcooliques. Ces produits sont indissociables de la production de biodiesel, qui utilise ces tourteaux. Face à l'image de nos routes désertées, nous pouvons imaginer l'inévitable dévalorisation

Afin de sécuriser la production d'huiles et protéines végétales et en soutien à la filière, il conviendrait d'instaurer, pour une durée limitée à six mois à compter de la fin des mesures de confinement, une réduction de la fiscalité applicable à ce biocarburant, qui, en outre, représente une solution d'avenir. La parole

Cela a été dit, l'effet cumulé de la faible demande en carburant, liée aux mesures de confinement mais également à la chute du prix du pétrole, a conduit à une baisse importante de la consommation de biodiesel. La perte de débouchés est de l'ordre de 75 %. la filière française a poursuivi sa production pendant la crise, afin de maintenir l'approvisionnement stratégique en tourteaux de colza, en huiles alimentaires, mais aussi en glycérine, matière première importante pour la production de gel hydroalcoolique. Cette situation a conduit à la constitution de stocks importants de biodiesel, que la filière aura des difficultés à valoriser. Une fois les mesures de déconfinement prononcées, cela déstabilisera durablement la filière ainsi, bien

pourtant utiles aux professionnels, ont été supprimées : le remboursement de 2 euros par hectolitre sur le gazole, dont bénéficiaient les poids lourds transportant des marchandises, et le tarif réduit de TICPE sur les carburants, sous condition d'emploi et sous réserve de quelques aménagements.

dit plusieurs fois aujourd'hui -ont augmenté et qui est touché au premier chef par les mesures de confinement. Le transport de marchandises poursuit son activité- là, pour le coup, il y a de l'activité -tout en étant sensiblement déstabilisé dans son organisation et affecté dans sa trésorerie. La plupart des chantiers navals sont à l'arrêt, du fait des mesures sanitaires, et pourraient pâtir d'une baisse durable des commandes, en particulier dans le domaine des activités de plaisance. il devient urgent de donner une suite à deux mesures adoptées par le Sénat mais non conservées dans le texte final de la loi de finances initiale. Il s'agit de revenir sur la suppression de remboursement de TICPE dont disposaient les poids lourds et d'appliquer aux activités de réparation navale le tarif réduit dont bénéficient les activités de manutention, ces activités étant très proches l'une de l'autre, tant par leur contenu que par leur localisation.

sur le gazole acquis en France accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l'activité de transport routier de marchandises. L'augmentation, L'augmentation, initialement prévue au 1 janvier 2020, ne prendra réellement effet qu'à compter du 1 juillet de la même année, les dépôts des dossiers de remboursement partiel de la TICPE du gazole n'intervenant qu'à échéance semestrielle. Toutefois, au regard de la crise liée au Covid-19 et de l'incertitude de la reprise, car le secteur lui-même de la reprise progressive des secteurs clients, le report de cette augmentation permettrait d'améliorer la trésorerie des entreprises de transport, aujourd'hui durement touchées par l'arrêt de leur activité. Les enquêtes conduites par les organisations professionnelles du transport routier démontrent clairement que les flux sont totalement désorganisés et que le transport se fait à perte ou sans réelle marge. Tous ces éléments ont été objectivés par le Comité national routier. La réalité est encore plus difficile pour le reste des entreprises, celles qui travaillent notamment pour l'industrie, les travaux publics ou encore l'automobile : 81 % d'entre elles sont en arrêt total ou en très forte baisse d'activité. En moyenne, les chefs d'entreprise estiment avoir perdu 48 % de chiffre d'affaires

en application des dispositions de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006. Cet amendement vise donc à soutenir les trésoreries exsangues des entreprises du transport routier de marchandises, car il est primordial de ne pas hypothéquer la reprise lente et progressive de l'économie en ne soutenant pas le maillon essentiel du transport et de la logistique, dont l'ensemble de l'économie de production, de distribution et de commerce aura besoin pour redémarrer au cours des prochains mois. Le coût de cette mesure est estimé à 210 millions d'euros dans sa globalité : 70 millions en 2020 et 140 millions en 2021. Quel

en compte l'ensemble des dépenses exceptionnelles liées à la mise en oeuvre des mesures spécifiques de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Cette épidémie a engendré des surcoûts particuliers pour les collectivités locales,

Concernant l'impôt sur le revenu, le prélèvement à la source mis en place par le gouvernement de François Hollande trouve ici une conséquence immédiate sur la perception contemporaine de l'impôt. On voit bien que cette baisse de l'impôt sur le revenu est adaptée à la situation.

celle de 54 millions d'euros de l'impôt sur la fortune immobilière, qui anticiperait une baisse de l'immobilier.

au remboursement accéléré de la TVA et au rattrapage du retard dans les services de la publicité foncière, qu'il conviendrait de ne pas oublier. Ce service public a subi de nombreuses suppressions d'emplois.